Ils représentent 4 % des élèves du primaire, 12 % des collégiens et de 2 % à 3 % des lycéens. Ce phénomène toucherait un élève sur dix et, parmi eux, 5 % subiraient un harcèlement sévère ou très sévère. Fait particulièrement inquiétant, le harcèlement scolaire peut intervenir très précocement puisque, selon l'UNICEF, 47 % des enfants en classe de cours préparatoire en font l'expérience. S'il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, le harcèlement à l'école prend cependant une ampleur inédite, plus continue et à plus grande échelle, avec l'avènement des réseaux sociaux et du cyber-harcèlement, qui touche particulièrement les filles. Par ailleurs, nous savons bien que la problématique du harcèlement, c'est l'isolement. Les enfants victimes ont trop souvent tendance à se replier sur eux-mêmes et à se sentir coupables. C'est précisément contre ce repli qu'il faut lutter, afin de permettre aux enfants victimes de trouver au sein de leur établissement scolaire un soutien et une écoute. Si l'éducation nationale a, sur son site internet, mis à disposition des outils à destination des enseignants afin qu'ils puissent mettre en place des actions préventives contre le harcèlement, rien n'est prévu dans leur formation pour leur permettre d'en détecter les signes et d'y répondre de manière adaptée.

prévu au sein des établissements pour recevoir les enfants victimes. Je le rappelle, les conséquences du harcèlement scolaire peuvent être dramatiques pour nos enfants et laisser des séquelles à vie, voire, dans les cas les plus extrêmes, mener au suicide. Aucun enfant ne devrait avoir peur d'aller à l'école. Il est indispensable que nos établissements scolaires puissent être des espaces où chaque élève apprend et grandit en sécurité. Très bien

mesures mises en place et les perspectives. Nous avons la volonté de ne pas laisser les victimes et leurs familles seules face à ce type de situation. L'école doit être avant tout le lieu de la confiance, du respect d'autrui et du bien-être. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a a une action centrale ; les académies, les écoles et les établissements sont mobilisés contre toutes les formes de harcèlement. Cette politique se décline selon quatre axes. Premièrement, il s'agit d'informer et de sensibiliser les élèves, les familles et l'ensemble des partenaires, afin d'interpeller et de mobiliser largement.

interviendra dans les prochains mois ; il s'agira bien évidemment de faire le point sur ce sujet et de voir les adaptations possibles. Quatrièmement, il s'agit de prendre en charge chaque situation, plus précocement et plus efficacement, par une professionnalisation des acteurs de terrain aidés des 310 référents académiques, la mobilisation des référents académiques et départementaux qui prennent contact avec la victime, sa famille et avec l'établissement concerné pour résoudre la situation, la mise en place dans chaque école et dans chaque établissement de protocoles de prise en charge et celle d'un numéro, le 30 20, dédié à l'écoute, au conseil et à l'aide aux victimes, aux familles, aux témoins et aux professionnels.

Le département de l'Orne accueille trois par trois des prisonniers en vue de les « déradicaliser », jusqu'à concurrence des quarante places créées. Aujourd'hui, les médecins du CPO interviennent dans les centres pénitentiaires de l'Orne auprès de prisonniers présentant des troubles du comportement avérés, pour lesquels il existe des thérapies ou des traitements médicamenteux appropriés. Or, jusqu'à preuve du contraire, la radicalisation comme l'intégrisme ne sont pas des maladies psychiatriques, d'où le questionnement légitime des médecins du CPO. Cette mesure déstabiliserait l'organisation médicale du CPO, aujourd'hui tendue à cause de la situation de la démographie médicale que nous connaissons tous, qui touche aussi fortement la médecine psychiatrique. De manière plus globale, la psychiatrisation, la pathologisation de la radicalisation est un véritable non-sens et montre que les sanctions éventuelles encourues par les personnes concernées ne sont pas du tout adaptées à la réalité de l'horreur de ce fléau.

Un quartier de prise en charge de la radicalisation, un QPR, a ouvert le 24 septembre 2018 au sein du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du plan national de prévention de la radicalisation annoncé le 23 février 2018 par le Premier ministre et constitue l'une des modalités de gestion des quelque 500 détenus actuellement incarcérés dans les prisons françaises françaises pour des faits de nature terroriste. Ces quartiers, qui s'inscrivent dans une stratégie nationale d'évaluation et gestion des détenus radicalisés, ont vocation à accueillir, après une évaluation pluridisciplinaire, les individus présentant un niveau de prosélytisme idéologique et d'incitation au passage à l'acte tel que nous ferions courir courir de grands risques au personnel pénitentiaire, aux partenaires intervenant en prison, mais aussi à la société tout entière, si nous les laissions en détention ordinaire au contact des détenus les plus vulnérables. Les QPR sont destinés non déradicaliser »- ce terme fait d'ailleurs débat dans le milieu académique -les détenus concernés, mais à permettre leur gestion très sécurisée et séparée du reste de la détention, tout en mettant en place une prise en charge globale, individuelle et collective, visant au désengagement de la violence et à la déconstruction de l'appareil idéologique d'une organisation terroriste qui a déjà, bien trop nombreuses reprises, frappé et endeuillé notre pays. L'intervention des personnels de santé au sein de ce quartier spécifique ne répond pas à une logique de psychiatrisation de la radicalisation. Elle s'inscrit dans le cadre général de l'accès aux soins des personnes détenues, tel que le définit la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, qui a posé le principe du transfert de la prise en charge sanitaire des personnes détenues au ministère chargé de la santé. Le centre psychothérapique de l'Orne intervient conformément à ces dispositions au sein du QPR de Condé-Sur-Sarthe, l'intervention des personnels du CPO, à l'instar d'ailleurs de celle des professionnels du centre hospitalier d'Alençon sur le volet somatique, s'effectuant dans le cadre général de la prise en charge de la santé mentale des détenus. Si ces professionnels prennent en charge un public spécifique, nous n'entendons pas pour autant « psychiatriser » la radicalisation, les personnes détenues inscrites dans un processus de radicalisation pouvant, comme toute personne placée sous main de justice, présenter des troubles mentaux, des troubles psychiatriques ou une souffrance psychique. Toutefois, la réponse au terrorisme ne peut être que collective et concertée : c'est tout le sens du plan national de prévention de la radicalisation que soutient l'ensemble du Gouvernement. La mobilisation de l'ensemble des professionnels intervenant auprès des détenus, qu'ils soient radicalisés ou non, est nécessaire, chacun devant oeuvrer dans son domaine de compétence et dans le respect du cadre prévu par la loi, mais de la façon la plus concertée possible. Nous savons, à cet égard- ce point est fondamental -, que les conditions de sécurité des personnels soignants font l'objet d'une attention toute particulière de l'administration pénitentiaire et d'échanges réguliers. Cette concertation locale et l'accompagnement des équipes sanitaires seront poursuivis et et accentués. Mme la garde des sceaux et Mme la ministre des solidarités et de la santé comprennent les légitimes inquiétudes des professionnels du centre psychothérapeutique de l'Orne. Les enjeux collectifs sont de taille : mettre en oeuvre une prise en charge globale du détenu radicalisé en prison et s'assurer de sa poursuite lorsque le détenu est libéré. Une instruction commune aux ministères de la justice et des solidarités et de la santé

Alors que l'année 2018 s'achève, seuls 60 000 contrats subventionnés ont été signés. Le faible nombre de demandes de contrats aidés est lié à la hausse du coût du dispositif et aux contraintes administratives grandissantes, qui découragent de nombreuses structures à y avoir recours, malgré des besoins importants. Ces contrats, qui ont vocation à permettre l'insertion de personnes éloignées du marché de l'emploi, sont essentiellement signés dans des zones où le chômage est plus élevé que la moyenne nationale. Dans la commune de Marans, en Charente-Maritime, le centre social Les Pictons employait en contrat aidé Celui-ci participait à l'engagement de jeunes en difficulté dans des associations sportives et culturelles ; il les amenait à une réelle prise de conscience de leur citoyenneté. Avec le remplacement du contrat aidé par le parcours emploi compétences, la prise en charge de cet emploi s'établit désormais à environ 50 % du salaire, contre 75 % auparavant. Le centre social n'est plus en mesure d'assumer le coût de cet emploi. Rien ne garantit que les collectivités locales auront la capacité financière de compenser cette baisse des moyens. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement entend-il mettre en place un statut dérogatoire pour les animateurs de prévention en centres sociaux, afin que ces derniers puissent continuer à bénéficier d'une prise en charge des contrats à hauteur de

Concrètement, les parcours emploi compétences, les PEC, comportent un accompagnement renforcé du bénéficiaire tout au long du contrat et une sélection des employeurs et des postes offrant les conditions d'un parcours insérant par la formation et le développement des compétences. À ce titre, les premiers résultats sont positifs les PEC sont plus ciblés sur les publics éloignés de l'emploi et les employeurs s'engagent davantage sur des formations qualifiantes ou permettant le développement de compétences identifiées. Concernant le taux de prise en charge, leur niveau élevé dans le passé n'a pas été un gage de qualité. Un taux de prise en charge spécifique n'est donc pas la solution. Le Gouvernement entend soutenir les structures associatives par d'autres moyens. J'ai présenté la semaine dernière la feuille de route pour le développement de la vie associative, qui comprend quinze mesures ambitieuses, notamment un fort soutien à l'emploi associatif l'affectation annuelle, pendant les quatre prochaines années, de 1 000 postes FONJEP

Sans aller jusqu'à la personnalisation, nous pourrions utiliser les numéros jugés intéressants ou demandés par les contribuables dans la suite alphanumérique du système SIV. Cette nouvelle option permettrait de satisfaire la demande de nombreux propriétaires de véhicules, mais aussi de constituer une recette parafiscale extrêmement intéressante pour l'État. Cette requête a été faite dès 2009 par la Fédération française des véhicules d'époque- sans succès, malheureusement, la principale objection étant la surcharge de travail pour les services des préfectures. depuis la fermeture des guichets départementaux, la gestion des cartes grises est possible directement par internet ; elle est plus généralement assurée par des professionnels indépendants collecteurs de la taxe. » pourrait être mise en place sur le même principe, avec une société chargée de la gestion de la clientèle, de la détermination de la pertinence des numéros protégés et de la collecte de cette nouvelle recette fiscale. Sa rétribution serait fixée selon un barème à définir. Ainsi, avec un investissement de départ minime et sans frais d'exploitation, une rentabilité significative serait rapidement atteinte. De plus, l'abandon du fichier national des immatriculations, dit FNI, à la fin de l'année 2020, au bénéfice du SIV, représente une réelle opportunité. Les collectionneurs de véhicules anciens seront dans l'obligation de procéder à un changement d'immatriculation, avec dans ce cas la possibilité de la personnaliser. Pas moins de vingt pays européens ont d'ores et déjà mis en place la possibilité d'obtenir contre paiement

Laurent Nunez, qui reçoivent ce matin les représentants des syndicats de policiers dans le contexte que nous connaissons. La personnalisation des plaques, telle que pratiquée à l'étranger, nécessiterait de revenir sur l'architecture réglementaire et technique du système d'immatriculation des véhicules, le SIV, qui a été mis en place en 2009 afin de délivrer un numéro d'immatriculation définitif suivant le véhicule, et non le titulaire du certificat d'immatriculation. Changer ce système d'immatriculation à vie du véhicule, plus simple et plus efficace contre les fraudes et trafics en tout genre, reviendrait à mettre en oeuvre une réforme profonde et coûteuse, alors que le ministère de l'intérieur est déjà engagé dans une vaste transformation des modalités de délivrance des certificats d'immatriculation pour simplifier leur demande et dématérialiser leur traitement. Dans ce cadre, d'importants travaux de consolidation technique et fonctionnelle sont en cours. Cela rend inopportun et risqué de procéder à de nouvelles transformations structurelles à court terme, alors que le SIV est aujourd'hui un système d'information stratégique pour la sécurité de nos concitoyens sur les routes, la lutte de nos forces de l'ordre contre le terrorisme et la criminalité liée aux véhicules, l'activité économique de nos filières automobiles. L'introduction d'une personnalisation des plaques d'immatriculation pourrait donc se révéler aujourd'hui contre-productive, quand le ministère s'applique à rendre plus efficace et plus simple le système de délivrance des certificats d'immatriculation. Toutefois, il nous faudra nous interroger à l'avenir sur l'opportunité d'une telle modification, lorsque le système d'immatriculation actuel arrivera en fin de vie et que sa numérotation nécessitera

souhaiter renforcer la présence de l'État à la frontière franco-espagnole, notamment dans le département des Pyrénées-Atlantiques, pour ainsi mieux maîtriser les flux migratoires. Les chiffres suivants ont été avancés : sur les 48 000 entrées irrégulières

Je note que ce jeu de chaises musicales au sud de l'Europe est une nouvelle illustration flagrante du fait que le sujet de la politique migratoire ne peut être traité à la seule échelle nationale. Lorsque les États de l'Union européenne ne se coordonnent pas, il en résulte un isolement de chacun des pays membres, qui appliquent des solutions unilatérales. Cela peut aussi provoquer des tensions évitables sur notre territoire national.

Par ailleurs, l'une des solutions envisagées pour gérer ces enjeux transfrontaliers est la mise en place d'un coordonnateur de la sécurité, chargé de faire le lien entre les autorités douanières françaises et espagnoles à la frontière.

Depuis le début de l'année 2018, plus de 54 000 arrivées irrégulières de migrants ont été recensées en Espagne, soit une augmentation de 123 % par rapport à l'année précédente. L'Espagne devient ainsi le premier point d'entrée en Europe. Policiers français et espagnols coopèrent quotidiennement pour faciliter la prise en charge par les autorités espagnoles des personnes faisant l'objet d'une mesure de non-admission. Des renforts de CRS ont également été déployés à la frontière et permettent la tenue de deux points de passage autorisés majeurs. L'administration assure par ailleurs, sous le contrôle du juge, le respect des droits des personnes qui font l'objet d'un contrôle aux fins de non-admission sur le territoire français. La durée de retenue des personnes ne peut excéder quatre heures. En outre, les personnes retenues le sont dans des bâtiments qui disposent de sanitaires et se voient remettre des bouteilles d'eau, conditions qui satisfont également aux exigences posées par le juge administratif. la sénatrice, un coordonnateur pour la frontière franco-espagnole sera prochainement nommé pour superviser ces opérations et assurer un contact permanent de haut niveau avec les autorités espagnoles. Cela nous permettra de renforcer notre coopération avec le Gouvernement espagnol sur des sujets d'intérêt commun aux frontières de l'Union européenne, comme le soutien aux garde-côtes marocains pour dissuader les départs dans le respect du droit. Lors de la rencontre du ministre de l'intérieur avec son homologue espagnol, le 12 novembre dernier, a été réaffirmée la nécessité de poursuivre une approche européenne globale et coordonnée pour répondre aux défis migratoires actuels, en agissant sur le plan tant international qu'interne. Lors du conseil européen du 6 décembre la France défendra ses positions afin de faire aboutir les négociations sur le régime européen de l'asile pour contenir les flux migratoires secondaires dans l'Union européenne et assurer une solidarité efficace ; le Président de la République est pleinement mobilisé sur ce sujet. Elle soutiendra

concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, du fait de la jurisprudence de la Cour de justice européenne. L'arrêt Matzak menace la pérennité du modèle français de secours. En effet, assimiler les sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs conduirait à appliquer au volontariat des règles de repos quotidien de sécurité et de plafond de temps de travail qui rendraient impossible à toute personne en activité de devenir sapeur-pompier volontaire. Ce serait la fin d'un modèle unique d'engagement citoyen altruiste et généreux, avec une ressource en sapeurs-pompiers volontaires considérablement réduite. Disons-le clairement : sans volontariat,

Disons-le tout aussi nettement, nous ne pouvons accepter que cette menace mette en péril et les ressources, et la sécurité civile, et la continuité de l'engagement de celles et de ceux qui agissent de manière altruiste au profit de leurs concitoyens.

très clair en faveur d'un volontariat reposant sur un modèle altruiste, véritable socle du modèle français de secours et de gestion des crises,

unique ne soit en aucun cas remis en cause ? Quelles démarches entendez-vous engager ? Je rappelle que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France estime nécessaire la mise en chantier

son organisation et son implantation territoriale cohérente, il permet aussi bien de faire face aux accidents du quotidien que d'affronter les crises exceptionnelles. Ce modèle, garant de la sécurité des Français au quotidien, doit être protégé et conforté.

harmonisés et protecteurs. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018, dit « arrêt Matzak », suscite une inquiétude chez les sapeurs-pompiers volontaires, qui craignent une remise en cause du modèle français de sécurité civile. En effet, l'assimilation sans aménagement du volontariat à un travail pourrait limiter sa compatibilité avec tout autre emploi salarié en ce que le cumul d'activités résultant de cette assimilation pourrait potentiellement conduire à un dépassement des plafonds, rendant le salarié inemployable à l'issue d'une période d'activité de sapeur-pompier volontaire. Dès lors, le Gouvernement, qui entend et partage la préoccupation des sapeurs-pompiers volontaires et des élus, a immédiatement fait part de sa volonté de protéger notre système de secours, qui repose précisément, pour sa plus grande part, sur l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires. Plusieurs pistes de travail sont envisagées en vue de protéger ce modèle du volontariat, au travers de la transposition de la directive, d'une part, afin d'en exploiter les larges facultés de dérogation,

le lancement d'une expérimentation de l'intégration des missions locales au sein de Pôle emploi, annoncé par voie de communiqué de presse cet été par le Premier ministre. Cette mesure, qui ne figurait pas dans le rapport initial du comité « action publique 2022 » et qui n'a fait l'objet d'aucune concertation, remet en cause le modèle des missions locales. Ces dispositifs, qui accueillent 1,5 million de jeunes chaque année, dont plus de 30 000 en Seine-Maritime, mon département, sont pilotés aujourd'hui par des élus locaux au profit de leur territoire, dans le cadre d'une gouvernance associant collectivités, services de l'État, partenaires économiques et sociaux et et personnes qualifiées. Les missions locales bénéficient ainsi d'un important maillage de proximité et du soutien des départements et des régions. L'accompagnement qu'elles offrent aux jeunes est marqué par une approche à la fois globale et personnalisée des problématiques qu'ils rencontrent. Il prend notamment en compte leurs freins psychosociaux, leurs difficultés économiques, mais aussi leurs problèmes de santé, de logement, de mobilité. Les missions locales participent au développement social local et à la lutte contre la pauvreté des jeunes. Elles travaillent par ailleurs d'ores et déjà en liaison avec Pôle emploi, dans le cadre d'une collaboration efficace et complémentaire. Ces dernières années, de nombreux rapports et audits réalisés par l'Inspection générale des affaires ont attesté que les missions locales constituent le réseau le plus performant pour l'accompagnement social et professionnel des jeunes, pour un coût inférieur à celui des autres organismes. La perspective d'une fusion des missions locales et de Pôle emploi suscite donc l'inquiétude des acteurs locaux, en ce qu'elle fait craindre un éloignement des jeunes le plus en difficulté et un creusement des inégalités territoriales. Monsieur le secrétaire d'État, dans quelle mesure ces expérimentations seront-elles effectivement laissées à l'initiative des acteurs locaux ? N'institueront-elles pas un nouveau mode de gouvernante imposé par les services de l'État et de Pôle emploi,

le plus en difficulté, il y a cependant un aspect que nous pouvons améliorer : l'efficacité des relations entre Pôle emploi, les missions locales et les Cap Emploi, qui s'occupent des personnes en situation de handicap. Si, aujourd'hui, ces organismes se parlent et partagent leurs informations, aller plus loin, afin de pouvoir conduire des parcours d'inclusion plus efficaces. Il s'agit de construire un patrimoine commun, de partager des systèmes d'information ou des offres d'emploi pour pouvoir être plus efficaces collectivement, des antennes permettant aux missions locales d'assurer un service de proximité. En effet, il ne suffit pas d'attendre que les demandeurs d'emploi ou les jeunes viennent ; il faut aussi aller au-devant d'eux. C'est un aspect que nous souhaitons et que nous pouvons améliorer. C'est pourquoi, de façon générale, le Gouvernement soutient toutes les démarches qui visent à coordonner les offres de services, à partager les informations et à rechercher les synergies. Ainsi, à la demande des collectivités locales et de leurs élus- et seulement à leur demande -, le rapprochement entre les missions locales et Pôle Emploi pourra être expérimenté, selon des formes qu'il leur appartient de trouver. Monsieur le sénateur, nous partageons le même objectif. Il faut que les missions locales continuent et amplifient leur action auprès des jeunes, qu'elles soient bien en phase avec les problématiques d'apprentissage, d'accès à la formation et d'emploi, pour permettre à ces jeunes d'accéder à un avenir. La parole

ce qui me semble être en contradiction avec l'ambition du Président de la République de multiplier par cinq l'accueil des jeunes dans le cadre du plan Pauvreté. Je souhaite donc que le Gouvernement ait une attitude bienveillante à l'égard des amendements que nous défendrons en vue de rétablir ces financements.

Ils n'habitent pas non plus dans les plus petites intercommunalités, de moins de 10 000 habitants, qui ont un régime dérogatoire. Ils habitent dans des intercommunalités rurales

du ministre de l'intérieur, qui reçoit ce matin les représentants des syndicats de policiers, dans le contexte que nous connaissons. Il m'a demandé de vous répondre à sa place. Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est reversé aux collectivités territoriales et aux groupements afin de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation routière. Logiquement, les collectivités territoriales bénéficiaires de ce reversement disposent donc des compétences leur permettant de mettre en oeuvre ces travaux. C'est pour cette raison que, hors de l'Île-de-France, ce produit est attribué aux communes, sauf si celles-ci appartiennent à un groupement auquel elles ont délégué la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement. Des seuils démographiques permettent en outre de garantir l'équité des modalités de répartition actuelles du produit des amendes de police. En effet, la part de ce produit revenant

direct du produit des amendes. Une attention particulière a également été portée aux communes rurales dans le cadre de la décentralisation du stationnement payant. La loi de finances rectificative de 2016 a prévu que, à partir de 2019, les enveloppes départementales allouées aux petites communes seraient au moins égales à la moyenne des sommes allouées au titre des trois derniers exercices. Les communes de moins de 10 000 habitants qui n'ont pas choisi de mettre en place le forfait post-stationnement se voient ainsi préservées des conséquences de la baisse des recettes des amendes de police. Le Gouvernement est toutefois conscient que les choix d'organisation locaux peuvent parfois aboutir à des répartitions sous-optimales du produit des amendes de police. Il est donc ouvert à une modification réglementaire

Avec 27 médecins pour 10 000 habitants, toutes spécialités confondues, le département de l'Oise est confronté à un phénomène de désertification médicale catastrophique. Or les réponses apportées à ce terrible constat manquent d'efficacité, de stabilité et de clarté.

Heureusement, les présidentes des départements de l'Oise et du Val-d'Oise se sont entendues dernièrement pour sauver un EHPAD à Méru, l'État n'en pouvant mais. En définitive, les acteurs de santé comme les patients sont confrontés au flou et à l'illisibilité de la carte hospitalière

Concernant plus particulièrement le projet de regroupement des accouchements sur le site de Senlis, proposé par la communauté médicale, il vise à améliorer la qualité et la sécurité des soins par rapport à la situation actuelle, au travers d'un parcours de soins mieux organisé et plus lisible. Pour ce faire, il est nécessaire de transférer la réanimation néonatale et les soins intensifs néonataux sur le site de Senlis. Ce projet de regroupement permet par ailleurs de conforter le recrutement médical dans toutes les composantes professionnelles concernées- anesthésie, gynécologie-obstétrique et pédiatrie -en diminuant l'effort de permanence de soins médicale qu'exige le fonctionnement de deux lieux de naissance. Ce projet a fait l'objet de nombreux échanges et la démocratie sanitaire a pu largement en débattre. Soyez Soyez assuré qu'une attention particulière a été portée au suivi obstétrical pré-et postnatal des femmes afin qu'il s'organise sur les deux sites. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient la décision prise par la communauté médicale et la direction du GHPSO de regrouper les deux maternités sur le site de Senlis,

Des mesures de protection des troupeaux ont été prises au détriment du pastoralisme, mais elles sont inadaptées si l'on en juge par la recrudescence d'attaques et le nombre d'animaux victimes. Je rappelle d'ailleurs que le plan national d'action 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage est loin de répondre aux besoins des territoires et aux attentes de la profession agricole. C'est pourquoi je souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre, sur le coût réel de la politique actuellement menée en faveur des espèces protégées. Je ne parle pas des 30 millions d'euros consacrés aux indemnités et aux mesures de protection visant à compenser les pertes directes, dont vous êtes comptable avec votre collègue le ministre de la transition écologique et solidaire écologique et solidaire : je souhaite connaître le coût réel de la prédation, lié, pour les éleveurs, au stress, au manque de sommeil qui conduit à la maladie, voire au suicide, pour les bergers, au temps passé à compter les cadavres ou à rassembler les troupeaux en perdition après une attaque,

J'appelle son attention sur un problème dont j'ai pris la mesure au cours des derniers mois. La Manche est un département grand producteur de chevaux. Il est même l'inventeur du cheval de selle français.

soit reconnu comme équivalant à un diplôme agricole, afin que nos éleveurs de chevaux, qui ne sont pas si différents de nos éleveurs de bovins ou de moutons, puissent bénéficier des aides agricoles à l'installation.

est accordée à tout détenteur d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel option « conduite et gestion de l'exploitation agricole » ou au brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole

et les qualifications professionnelles délivrées par la Fédération française d'équitation ne visent pas l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole et ne confèrent donc pas d'emblée la CPA. Néanmoins, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et le ministère des sports accordent réciproquement des équivalences dans les enseignements généraux et/ou professionnels de leurs diplômes respectifs. Ainsi, afin de faire valoir ces

Pour obtenir la CPA, il lui restera à valider le ou les blocs de compétences manquants, par exemple celui portant sur la gestion comptable d'entreprise. Sous ces réserves, il doit être possible que l'équivalence soit reconnue.

et sept secondes. C'est précisément parce que nos jeunes diplômés de la filière équine se heurtent à des difficultés pour l'application de ces règles que j'ai posé ma question. Il me semble qu'un travail commun entre la filière équine

d'eau. Le même constat vaut pour les plantes intermédiaires, les surfaces d'intérêt écologique et ce que l'on nomme communément les « pièges à nitrates », ces cultures rendues obligatoires par l'Europe. C'est ainsi que, en plus de la sécheresse, les agriculteurs sont surveillés par l'administration qui, par ses contrôles obligatoires au constate des défauts de cultures dus à l'absence de pousse, susceptibles d'engendrer des pénalités ! Cet aléa climatique fait suite à quatre années de difficultés liées à la météorologie et à des cours mondiaux très bas. Alors que l'Allemagne a mis en oeuvre des plans d'urgence et que de nombreux pays ont obtenu de Bruxelles des dérogations pour les surfaces d'intérêt écologique, seule la France a demandé à ses agriculteurs d'effectuer des dépenses inutiles inutiles en semant malgré la canicule. L'Allemagne a très vite débloqué 340 millions d'euros pour ses agriculteurs, si bien que ceux-ci achètent aujourd'hui le fourrage qui nous manquera cet hiver

L'ensemble de ces mesures, sans comparaison avec ce qui a été mis en place dans les autres pays européens touchés par cette sécheresse, représente un apport de trésorerie exceptionnel pour les exploitants et des souplesses administratives leur permettant d'anticiper l'hiver et d'acheter les compléments nécessaires à l'alimentation des cheptels.

Faute d'entretien, ces bâtiments se dégradent et deviennent dangereux pour les occupants, les voisins ou les habitants de la commune. Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement susceptibles de causer un danger pour la sécurité des occupants, il notifie au propriétaire qu'une procédure de péril ordinaire va être engagée. Aux termes des articles L. 511-1 à L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité. Mais les petites communes n'ont plus les moyens de se substituer aux propriétaires défaillants. Dans certains cas, elles n'ont même plus les moyens de supporter les frais de contentieux. Lorsque Mme la ministre Jacqueline Gourault est venue assister à l'assemblée générale des maires du Jura, trois maires se sont ouverts à elle de leurs difficultés, et elle a évoqué l'idée de créer un fonds spécial dédié à cette problématique.

Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine, le maire peut en effet prescrire la réparation ou la destruction de bâtiments et mettre en demeure un propriétaire, par un arrêté de péril et à l'issue d'une procédure contradictoire, de prendre les mesures nécessaires. l'ANAH, peut accorder des subventions aux propriétaires pour financer la réalisation de travaux dans le cadre d'une procédure de police administrative de lutte contre l'habitat indigne. Lorsque les travaux ne sont pas réalisés par le propriétaire dans le délai qui lui est imparti, le maire a la possibilité de faire procéder d'office à leur exécution. Ces travaux sont alors réalisés pour le compte du propriétaire défaillant et à ses frais. Les communes peuvent en effet recouvrer les frais qu'elles ont avancés mais qui restent dus par le propriétaire défaillant. Le Gouvernement n'envisage pas de créer un fonds spécifique, madame la sénatrice. Toutefois, les maires ne sont pas seuls et l'État, avec ses opérateurs, apporte un soutien financier important aux opérations qu'ils mènent pour résorber l'habitat indigne. l'ANAH subventionne les travaux d'office réalisés par les communes au titre de diverses procédures, et cette subvention reste acquise à la commune, même après recouvrement complet des sommes engagées auprès du propriétaire. Même si le problème concerne un immeuble en copropriété, l'ANAH est en mesure de subventionner les travaux d'office décidés par le maire en substitution aux copropriétaires défaillants, qui ne paieraient pas leur quote-part de travaux. Lorsque l'action de la commune nécessite de prendre possession de l'immeuble du fait de l'inaction de son propriétaire, l'ANAH pourra désormais financer avec la collectivité ce type d'opération. Nous avons ainsi prévu, dans le PLF pour 2019, un budget de 15 millions d'euros à ce titre. Très récemment enfin, la loi ÉLAN est venue renforcer les moyens financiers dont disposent les collectivités territoriales pour mieux lutter contre ces situations d'habitat indigne. Elle leur transfère le bénéfice des astreintes imposées aux propriétaires indélicats pour que les travaux soient faits.

était enfin abandonné. Nous avons exprimé notre gratitude à Mme Jacqueline Gourault. Avec le président du conseil départemental du Nord, Jean-René Lecerf, nous nous sommes opposés à cette idée baroque d'un partage du territoire nordiste en trois entités distinctes, qui aurait créé un département-métropole fusionné au centre du territoire et deux super-arrondissements regroupant la Flandre intérieure et la Flandre maritime, d'une part, le Douaisis, le Valenciennois, le Cambrésis et l'Avesnois, d'autre part. Au-delà de l'ineptie géographique évidente, qui pouvait s'apparenter au partage de l'empire carolingien en 843 par le traité de Verdun entre les trois héritiers de Charlemagne, ce projet de fusion dénaturait complètement les équilibres sociaux, économiques et démographiques, dans un territoire déjà en forte souffrance sociale. Cette chimère de la fusion entre le département du Nord et la métropole européenne de Lille étant écartée, il ne faut cependant pas oublier les difficultés structurelles du département du Nord,

de relancer un vrai débat constructif avec les territoires sur la question de la nécessaire réévaluation de la participation de l'État aux aides individuelles sociales,

peine. Comment le Gouvernement envisage-t-il de remettre au centre des discussions avec les territoires la question de la péréquation nationale et d'une plus juste solidarité entre l'État et les territoires, d'une part, et entre territoires riches et territoires pauvres, d'autre

Les travaux menés par la mission dirigée par Alain Richard et Dominique Bur avaient pour but de trouver des solutions pour assurer une meilleure maîtrise de l'évolution des dépenses liées aux AIS et établir un équilibre financier pérenne. Le Gouvernement est pleinement conscient de la très forte croissance de ces dépenses au cours des dernières années, qui a conduit à la mobilisation de quatre fonds exceptionnels de soutien aux départements, instaurés dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2010, 2012, 2015 et 2016. Un fonds exceptionnel doté de 100 millions d'euros a été créé par la loi de finances rectificative pour 2017 afin de soutenir les départements confrontés aux situations financières les plus dégradées. À l'instar d'autres départements, le département du Nord a bénéficié d'aides exceptionnelles au titre de ces fonds : près de 55 millions d'euros lui ont été versés depuis 2013. Déterminé à aider les départements les plus exposés, le Gouvernement a également déposé un amendement au projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Cet amendement vise à créer un fonds de stabilisation doté de 115 millions d'euros sur trois ans pour accompagner dès 2019 une trentaine de départements présentant une situation financière dégradée et des restes à charge au titre des AIS supérieurs à la moyenne nationale. renforcer la péréquation horizontale des recettes des droits de mutation à titre onéreux, à hauteur de 250 millions d'euros dès 2019. Le Gouvernement examine attentivement la proposition de répartition faite par l'Assemblée des départements de France, du PLF pour 2019. Parallèlement à ces mesures, le Président de la République a présenté, le 13 septembre dernier, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Des financements seront ainsi apportés aux départements volontaires afin d'accompagner la dynamique de leurs dépenses en matière d'accompagnement social : 135 millions d'euros en 2019, 177 millions d'euros conscient des difficultés liées l'accueil des mineurs non accompagnés, le Gouvernement a également confirmé qu'un soutien financier renforcé, à hauteur de 141 millions d'euros en 2019, serait apporté aux départements, au titre tant de la phase en amont de la reconnaissance de la minorité que de la phase aval au titre de l'aide sociale à l'enfance. La parole

pour les populations vulnérables, des températures hivernales. Le plan prévoit différents niveaux opérationnels en fonction des températures ressenties lors des vagues de froid. Que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, les communes, quelle que soit leur taille, se mobilisent dans le cadre du plan Grand Froid. Cette mobilisation se traduit par la mise à disposition de locaux, la gestion de centres d'hébergement d'urgence ou encore la réservation d'appartements. Chaque année, l'État consacre plusieurs centaines de millions d'euros à la politique d'hébergement d'urgence. Pourtant, malgré ces dotations, dans des villes moyennes, périphériques comme Fécamp, en Seine-Maritime, la mise en oeuvre du plan s'avère très difficile. En effet, cette ville ne dispose pas d'un parc hôtelier ou d'un nombre de logements suffisants pour mettre à disposition des nuitées ou des logements en urgence. En outre, si le dispositif du 115 couvre les grandes villes avoisinantes, comme Le Havre, il ne concerne pas une ville périphérique comme Fécamp. Cette situation paradoxale est renforcée par l'absence de transports publics en soirée et la nuit. Ainsi, la commune doit se débrouiller pour aider des associations qui se mobilisent pour les personnes identifiées comme ayant besoin d'une solution d'hébergement d'urgence. Chaque situation est traitée au mieux, en mettant en oeuvre des solutions souvent bricolées et plus ou moins pérennes.

par la mise à disposition de locaux ou d'équipements. Je voudrais rappeler, même s'il ne s'agit pas d'un, que jamais aucun gouvernement n'a fait autant en matière d'hébergement. L'État finance et gère avec les associations 136 000 places pérennes ouvertes tout au long de l'année pour l'accueil des personnes sans domicile. Le Gouvernement a pérennisé 5 000 places d'hébergement d'urgence à la sortie de l'hiver dernier. Le budget de l'hébergement d'urgence sera une nouvelle fois en hausse en 2019, et nous avons préparé cet hiver très en amont avec un plan d'action, en lien avec les associations, les services de l'État et les collectivités. Julien Denormandie et Jacqueline Gourault ont réuni les associations à deux reprises, le 19 octobre et le 23 novembre derniers, afin de leur présenter le plan et d'échanger. Ils les réuniront chaque mois. À ce jour, le nombre de places mobilisables est d'ores et déjà supérieur de près de 8 000 à ce qu'il était l'année dernière. S'agissant de la veille sociale, dont relèvent les services du 115, les crédits qui lui sont alloués ont progressé de 40,5 % entre 2016 et 2018. En 2019, plus de 139 millions d'euros y seront consacrés, soit une progression de 5,9 % par rapport à 2018. S'agissant particulièrement des maraudes, 5 millions d'euros supplémentaires sont prévus en 2019, 1,2 million d'euros ayant déjà été notifiés aux services pour la période hivernale, dont 427 000 euros délégués en novembre 2018 pour que les maraudes puissent être renforcées dès cette année. Sur la base d'une enquête réalisée en octobre auprès des services de l'État, ces crédits ont pu être notifiés dans l'ensemble des régions métropolitaines, dont la Normandie, à hauteur de 76 000 euros, et dans de nombreux départements. De manière générale, le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que la politique d'accès au logement des personnes défavorisées soit fondée sur une analyse locale des besoins des territoires, particulièrement ceux des villes petites et moyennes. C'est la raison pour laquelle la loi ÉLAN, qui qui vient d'être publiée, prévoit notamment que le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées sera désormais opposable pour la délivrance des autorisations d'activité des centres d'hébergement et de réinsertion sociale,

de l'Europe et des affaires étrangères. Depuis les annonces du Premier ministre, le 23 février dernier, il est question qu'une délégation de service public, Business France, soit opérée par certaines chambres de commerce et d'industrie à l'étranger pour l'accompagnement de nos PME à l'international.

Selon la cartographie du printemps 2018, Business France a déjà quitté la Russie, Hong Kong, le Japon et l'Espagne, et doit se retirer de la Belgique, de Singapour, de la Norvège et des Philippines d'ici à la fin de

ont actuellement pour mission d'aider les entreprises françaises à trouver des débouchés dans leurs pays d'accueil. Elles accompagnent et conseillent les entreprises à toutes les étapes de leur développement. Plus largement, elles contribuent au rayonnement économique des territoires à travers un vaste plan d'action.

promouvoir l'attractivité du territoire national et les investissements étrangers, et de mettre en oeuvre une stratégie de communication et d'influence visant à développer l'image économique de la France à l'international. Avec des rôles quelque peu différents, comment imaginer que ces CCI, associations de droit local, se substituent à une agence de l'État, financée sur fonds publics à hauteur d'environ 200 millions d'euros chaque année ?

Le 23 février 2018 dernier, le Premier ministre a annoncé la stratégie du Gouvernement en matière de commerce extérieur. La réforme de notre dispositif de soutien public a pour objectif de rendre l'accompagnement de nos entreprises à l'export plus simple et plus accessible, notamment pour les PME et les ETI, Cette réforme s'appuie sur la coopération de l'ensemble des acteurs au sein d'un dispositif unifié, la « Team France export », et s'appuie sur deux piliers : la création de guichets uniques dans toutes les régions et une refonte du réseau des bureaux de Business France à l'étranger. La mise en place dans les régions de « guichets uniques » pour l'accompagnement à l'export repose sur la signature de conventions entre Business France et les CCI régionales. Dans ce cadre, Business France redéploie des effectifs au sein des CCI afin de renforcer leurs capacités de prospection et le suivi des entreprises exportatrices. Les CCI pourront ainsi bénéficier des compétences des collaborateurs de Business France. À l'étranger, l'équipe de l'export prendra la forme de guichets uniques, reposant sur la désignation de « correspondants uniques ». Ces derniers pourront être soit Business France en propre, soit, dans le cas d'un retrait de Business France, des opérateurs privés désignés après des procédures transparentes d'appel d'offres dans le cadre de concessions de service public ou de marché public de services. Le Premier ministre a cité, le 23 février dernier, huit pays susceptibles de faire l'objet d'une expérimentation visant à confier l'accompagnement des entreprises à un opérateur privé. Dans ces huit pays- la Russie, la Belgique, la Norvège, la Hongrie, le Maroc, les Philippines, Singapour, le Japon et Hong Kong -, le Gouvernement a fait le choix de mener une expérimentation de retrait de Business France, qui concernera la totalité ou une partie de l'activité de l'opérateur.

Comme dans le cas du dispositif déployé sur le territoire national, il s'agit donc non pas d'arrêter un schéma identique dans tous les pays, mais de proposer un accompagnement adapté aux différentes situations économiques et commerciales, l'opérateur veillant à garantir une qualité de services homogène. Une concession de service public sera mise en place au 1 janvier 2019 dans six pays : la Belgique, la Norvège, la Hongrie, le Maroc, les Philippines et Singapour. La procédure d'appel d'offres publique visant à désigner un concessionnaire, qui peut être une chambre de commerce à l'étranger ou tout autre acteur privé, arrive à son terme. Les vainqueurs des appels d'offres seront désignés cette semaine. Au Japon et à Hong Kong, Business France a eu recours à un marché public de services pour sélectionner un prestataire exclusif. Les deux chambres de commerce françaises qui ont été choisies réaliseront cette prestation.

M. le ministre de l'économie et des finances. Il existe aujourd'hui dix-huit zones touristiques internationales- ZTI -sur l'ensemble de la France, dont douze à Paris intra-muros. Celle du 17 arrondissement- mon arrondissement d'élection -aurait pu disparaître en début d'année, mais la bonne collaboration entre le maire de l'arrondissement, Geoffroy Boulard,

ont la possibilité d'ouvrir le dimanche et en soirée toute l'année, en vertu d'accords signés avec les salariés. Avec deux ans de recul, la chambre de commerce et d'industrie de Paris a publié, cette année, une étude sur l'impact de la création de ces zones privilégiées dans la capitale. Le résultat est sans appel : l'ouverture des commerces le dimanche dans les ZTI est un succès. La fréquentation des lieux est en hausse de 20 % et l'ouverture dominicale a déjà permis aux grands magasins de la capitale d'augmenter leur chiffre d'affaires d'environ 10 % et de créer 1 000 emplois. Paris est la première destination touristique mondiale, mais rien n'est jamais acquis. Paris est une ville monde, en concurrence avec Londres, Berlin, Rome ou New York, et l'ouverture des commerces le dimanche s'inscrit dans une tendance mondiale. Aussi, comme le préconise un très récent rapport parlementaire rendu par nos collègues députés Philippe Huppé et Daniel Fasquelle, pourquoi ne pas créer une zone touristique internationale unique sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris, notamment pour éviter les effets de bord sur les baux commerciaux inhérents au zonage

Le Gouvernement a pleinement conscience du rôle de la ville de Paris pour l'attractivité touristique et l'activité économique. S'agissant de l'évolution du nombre de commerces ouverts à Paris le dimanche dans les zones touristiques internationales, les données sont publiées sur le site de l'observatoire des commerces dans les zones touristiques internationales, créé par arrêté interministériel du 20 juin 2016. Entre septembre 2015 et février 2017, une hausse très significative, de 62 %, du nombre de commerces ouverts le dimanche dans les ZTI a été observée. La chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France a effectivement proposé de faire de l'ensemble de la ville de Paris une zone touristique internationale. Cette proposition a été expertisée de manière approfondie. Il s'avère que la création d'une telle zone pourrait créer une rupture d'égalité entre les commerçants parisiens et ceux du reste de la France. Une telle rupture d'égalité semble difficilement justifiable. En outre, en l'état du droit, la ville de Paris dans son ensemble ne peut répondre aux critères d'une zone touristique internationale. En effet, la totalité des quartiers de Paris intra-muros ne présente pas un rayonnement international, une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France- ce sont là les trois critères permettant de définir une ZTI. Accéder à cette demande reviendrait donc à remettre en cause la politique actuelle de zonage s'appliquant pour l'ouverture dominicale des commerces, qui repose sur des critères fixés par la loi. Enfin, un bilan économique des zones touristiques internationales créées en application de la loi du 6 août 2015 sera présenté au Parlement début 2019. Sur cette base, l'opportunité d'améliorer ou de simplifier le régime des ZTI pourra être examinée. C'est peut-être alors que des réponses plus propres à vous satisfaire, madame la sénatrice, pourront être apportées

Monsieur le secrétaire d'État, le transfert au secteur privé de la société Aéroports de Paris, ou ADP, prévu dans le projet de loi PACTE fait l'objet de nombreuses oppositions, à droite comme à gauche.

sens, c'est une vue de court terme qui sacrifie sans états d'âme une part du patrimoine de l'État. Dans mon département, le Val-de-Marne, les inquiétudes et la mobilisation sont fortes quant aux conséquences de cette privatisation. Conséquences sur l'emploi tout d'abord : plus de 28 plus de 28 000 personnes travaillent sur le site d'Orly, dans un bassin économique de plus de 157 000 salariés, qui comprend également le marché international de Rungis. Conséquences sur l'environnement comment comptez-vous faire prévaloir les intérêts environnementaux des populations sur les intérêts économiques d'un concessionnaire privé qui, à n'en pas douter, remettra en cause les dispositifs de limitation des mouvements et le couvre-feu ? De plus, l'arrivée d'investisseurs privés majoritaires au sein du capital d'ADP risque de remettre en cause l'ensemble des stratégies territoriales défendues par les collectivités locales et l'État dans le cadre du projet du Grand Paris Express et de tous les schémas d'aménagement. Enfin, faut-il rappeler que les aéroports de Paris constituent la première porte d'entrée sur le territoire et, à ce titre, garantissent à la fois la sûreté nationale et la sécurité intérieure ? Monsieur le secrétaire d'État, au regard de tels enjeux,

secrétaire d'État. Madame la sénatrice Cohen vous avez appelé l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, retenu aujourd'hui, sur le processus de privatisation du groupe ADP. Je souhaite vous apporter en son nom les éléments de réponse suivants. Le projet de loi autorisant la privatisation d'ADP tient compte des enjeux pour les usagers et les territoires. Il prévoit des dispositions pour renforcer les leviers de régulation et de réglementation en matière de qualité de service, de sécurité, d'impact environnemental et d'intégration dans les territoires.

L'État pourra également imposer à l'opérateur de maintenir une qualité de service aux meilleurs standards des aéroports internationaux. S'agissant des employés d'ADP, le projet de loi PACTE précise que la privatisation n'a pas d'impact sur les statuts du personnel. La modification de ces statuts reste soumise à l'approbation de l'État. La protection des communes riveraines contre les nuisances sonores et de la qualité de l'air ne sera pas altérée par la privatisation : les normes aujourd'hui en vigueur, qu'elles soient législatives ou réglementaires, devront être appliquées par ADP, quel que soit son actionnariat, notamment celles instaurant un couvre-feu entre 23 heures 30 et 6 heures du matin ou le plafond du nombre de créneaux horaires attribuables annuellement à Orly. Afin de garantir les meilleures conditions de concertation avec les collectivités territoriales et les associations de riverains,

sur le nécessaire respect des dispositions légales en vigueur, s'agissant de la souscription des contrats d'assurance

que les contrats d'assurance obsèques sont très encadrés, notamment par l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales.

cet article, « toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite ».

Cependant, la loi doit être appliquée dans son intégralité. Dans la mesure où les signalements que vous nous faites ne nous sont pas connus de manière suffisamment précise pour que nous puissions vous apporter une réponse technique à ce stade, le ministère de l'économie et des finances souhaiterait pouvoir continuer à travailler avec vous sur la base

et les transporteurs, dont le bilan est déjà souvent dans le rouge malgré le taux réduit de TICPE. La transition énergétique doit être raisonnée, c'est-à-dire qu'elle doit permettre la poursuite de l'activité économique, notamment en milieu rural. Monsieur le secrétaire d'État, écoutez, entendez l'angoisse des Français les moins favorisés

vous nous interrogez sur la hausse de la fiscalité sur les carburants. Je tiens à souligner que l'engagement de l'économie nationale dans la transition énergétique doit rester une priorité, dont la mise en oeuvre est notamment assurée par la hausse progressive, décidée il y a plusieurs années, Cette transition doit être accompagnée afin de ne pas obérer le pouvoir d'achat de nos concitoyens en période de forte hausse. Ainsi, dans son discours pour l'installation du Haut conseil pour le climat, le Président de la République a souhaité que soit mise sur pied une méthode sur la base d'un rendez-vous trimestriel, permettant d'adapter les nouvelles hausses de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'évolution des marchés internationaux du pétrole dans le cas d'une envolée des prix, cela afin d'en atténuer les effets. Le Gouvernement a ainsi engagé des travaux pour aboutir rapidement à un système efficace et robuste, qui sera soumis au Parlement d'ici à la fin de l'année dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances. Il convient aussi de rappeler que des mesures spécifiques existent d'ores et déjà en faveur du monde rural. Ainsi, les consommations de carburant pour les transports collectifs ne subissent pas la hausse programmée sur le quinquennat. La consommation de carburant par le secteur agricole continuera à bénéficier d'un tarif très réduit, nonobstant la remise en cause du tarif du gazole non routier et sachant que la procédure de remboursement de taxe va être remplacée par l'application d'un tarif réduit appliqué directement à la pompe. Ce sont ainsi 480 millions d'euros de trésorerie annuelle qui seront restitués au secteur agricole.

Nous avons aussi pris la décision d'élargir le bénéfice du chèque-énergie, de manière à mieux aider les ménages les plus modestes ; cela concernera plusieurs millions de ménages. Monsieur le sénateur, le

de l'usine et du pôle de recherche et développement situés à Fondettes, dans l'Indre-et-Loire, et, par voie de conséquence, le licenciement imminent de ses 161 salariés. Cette fermeture touche un territoire qui a déjà subi les restructurations de Michelin en 2014 et de Tupperware en 2017. Un plan de sauvegarde économique a été lancé. Il concerne 130 employés de l'usine de production et les 16 salariés du centre de recherche et de développement, tandis que 14 employés devraient se voir proposer un transfert vers le site de production d'Orléans. Ce sont donc 161 salariés et leurs familles, installés dans toutes les communes de la métropole tourangelle, qui sont aujourd'hui inquiets pour leur avenir. Les premières lettres de licenciement devraient arriver au mois de mai 2019. L'entreprise explique la fermeture de l'usine par sa surcapacité de production. La décision de fermer le site de Fondettes est cependant difficilement acceptable pour les employés comme pour les élus. Le groupe suédois est, en effet, dans une situation économique et financière favorable, avec un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros en 2017.

Spécialisés dans la fabrication de plaquettes pour l'industrie automobile, les employés de Sandvik ont des compétences pointues dans un domaine très spécifique. Si nous ne pouvons agir sur le choix de cette entreprise d'abandonner l'usine située à Fondettes, il s'agit désormais de trouver rapidement un repreneur. Ce repreneur devra être capable de valoriser et de maintenir l'expertise des personnels industriels et de recherche. Si les salariés de l'usine venaient à être licenciés, ils auraient du mal à trouver un nouvel emploi en raison de la spécificité de leur métier, mais aussi de leur moyenne d'âge élevée. Le Gouvernement, qui considère que le maintien de l'activité de cette usine relève de l'intérêt national et territorial, a enjoint à la société Sandvik de trouver un repreneur sérieux. Or, enjoindre ne suffit pas, il faut aussi s'assurer du sérieux et de l'effectivité des démarches engagées par Sandvik. Il s'agit pour l'État d'oeuvrer pour qu'un repreneur puisse être trouvé rapidement. Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour préserver l'outil de travail et le savoir-faire unique des salariés de cette usine ? Comment compte-t-il accompagner la société Sandvik dans ses démarches ? La parole

Le groupe Sandvik a en effet annoncé le mois dernier la fermeture de son site de Fondettes et, par voie de conséquence, la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi touchant 130 employés de l'usine de production et 16 personnes du centre de recherche et développement, 14 autres salariés devant être transférés sur le site d'Orléans.

Comme vous le rappelez, le personnel de cette usine qui produit des outils d'usinage de haute technicité est très qualifié. Dès lors, nous concentrons tous nos efforts, en étroite association avec la métropole et les autres acteurs du territoire, sur la recherche d'un repreneur industriel. S'il ne nous appartient pas de juger et d'empêcher la réorganisation de Sandvik, nous ne laisserons pas ce grand groupe, qui réalise 8,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une marge opérationnelle que l'on peut qualifier de très confortable, ne pas consacrer tous les moyens à sa disposition à la recherche active d'un repreneur, sur une durée suffisamment longue pour que cette recherche puisse aboutir. C'est ce que les services du ministère ont signifié de façon très ferme aux dirigeants de l'entreprise, qu'ils ont reçus à Bercy. Nous avons déjà obtenu que Sandvik établisse et diffuse une liste des machines qui pourraient rester sur site et intéresser d'éventuels repreneurs. Un cabinet a également été mandaté par le groupe pour la recherche de repreneurs.

Le maintien de l'unité de recherche et de ce laboratoire est une priorité absolue du Gouvernement, et nous appelons Sandvik à prendre toutes ses responsabilités sur ce sujet essentiel. Vous l'aurez Vous l'aurez compris, le Gouvernement est mobilisé pour permettre le maintien d'une activité industrielle et d'une capacité de recherche et développement de haut niveau sur le site de Fondettes, et ce de façon pérenne. Nous comptons beaucoup

à la commande publique. Malheureusement, le projet d'élaboration de ce nouveau code semble se restreindre à une simple rationalisation des textes encadrant des dispositifs existants. Pour trois mesures qui ne sont pas mineures sont à noter : le relèvement du taux minimal du montant des avances, la diminution du montant de la retenue de garantie et la réduction des retards de paiement. Monsieur le secrétaire Quand on se déplace sur le terrain et que l'on prend le temps d'écouter ceux qui préparent les marchés publics et ceux qui y répondent ou souhaiteraient y répondre, on constate de lourdes rigidités, voire des blocages insurmontables. Ces obstacles vont à l'encontre des attentes de nos citoyens

accessible à tous fixe désormais un objectif de 50 % de produits locaux ou de qualité servis en restauration collective, dont 20 % de bio. Pourquoi ne pas saisir l'occasion de la création de ce code code de la commande publique pour marquer notre soutien à une transition écologique orientée vers les circuits courts et un approvisionnement local des organismes de restauration collective, comme cela a été réclamé durant les états généraux de l'alimentation

Lorsque les marchés existent et que l'allotissement fonctionne, il faut s'assurer que les opérateurs locaux ont connaissance de ces marchés et les aider à se structurer pour qu'ils soient en mesure d'y répondre. Il est temps que la commande publique favorise l'adoption d'une logique de projet territorialisée pour véritablement se faire l'outil de nos politiques de progrès social et environnemental. Monsieur le secrétaire d'État, allez-vous permettre aux PME agricoles de proximité d'accéder plus facilement aux marchés publics, dès la création de ce nouveau code de la commande publique ? Il serait dommage de manquer ce rendez-vous !

Les réformes visant à rendre la commande publique plus simple et plus attractive pour les PME sont donc portées par d'autres vecteurs législatifs et réglementaires. Leurs dispositions seront néanmoins consolidées le moment venu dans le code de la commande publique qui entrera en vigueur le 1 avril 2019. Ces réformes comportent des mesures concrètes pour les acheteurs publics comme pour les entreprises. Il s'agit notamment de l'augmentation de 5 % à 20 % du montant des avances forfaitaires versées aux titulaires des marchés publics de l'État, de la diminution de 5 % à 3 % du taux de retenue de garantie lorsqu'elle doit être constituée dans les marchés de travaux, l'obligation de prévoir des prix révisables, pour éviter de faire supporter par les fournisseurs les aléas majeurs des conditions économiques, comme c'est le cas pour les matières agricoles, et enfin de l'interdiction de la pratique des ordres de service à zéro euro, qui conduisait certaines collectivités à faire supporter des charges supplémentaires à leurs prestataires de travaux publics. En matière d'accès des PME nationales à la commande publique, l'attribution des marchés publics sur la base d'un critère de préférence locale se heurterait aussi bien à la Constitution qu'au droit européen. Par sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel affirmé que la liberté d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats à des contrats de la commande publique étaient des principes à valeur constitutionnelle découlant des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur les critères de choix dans les marchés publics et a constamment réaffirmé l'interdiction des critères visant à réserver les marchés publics à des opérateurs économiques installés dans un ressort géographique donné et des critères relatifs à l'utilisation de produits locaux. de tels critères porteraient atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité ou de non-discrimination. Ces principes s'appliquent aussi pour les entreprises de pays tiers à l'Union européenne, mais signataires, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, de l'accord « marchés publics Pour autant, le droit de la commande publique ne fait aucunement obstacle à la mise en oeuvre d'une politique responsable d'achats alimentaires visant à l'emploi de produits de qualité, segment sur lequel nos agriculteurs sont particulièrement bien placés. L'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pose une obligation de principe d'allotir les marchés publics afin de faciliter l'accès des PME à la commande publique. Un allotissement fin, notamment par type de denrée et par territoire, permet de susciter une large concurrence et de lever les obstacles à l'accès à la commande publique des producteurs locaux et de leurs groupements. Les articles 30 et 38 de la même ordonnance font obligation aux acheteurs, lorsqu'ils définissent leurs besoins, de prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, et autorisent la prise en compte de ces considérations dans les conditions d'exécution d'un marché public, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché. Les acheteurs publics peuvent ainsi exiger que les fournisseurs garantissent la fraîcheur et la saisonnalité de leurs produits. De même, les conditions d'exécution peuvent inclure des exigences en matière de sécurité et de célérité des approvisionnements alimentaires. Les acheteurs peuvent également recourir aux spécifications techniques définies par référence à des labels permettant de garantir la qualité des produits et de leur production, comme ceux ayant trait aux « spécialités traditionnelles garanties » ou à l'agriculture biologique, en vertu de l'article 10 du décret du 25 mars 2016. La qualité des offres peut s'apprécier au regard de l'effort de réduction des transports, dès lors que celui-ci a, par exemple, pour effet de limiter l'émission de gaz à effet de serre. La rapidité d'intervention d'un prestataire, ainsi que les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture sont, aux termes de l'article 62 du décret relatif aux marchés publics, des critères de choix autorisés, pour autant qu'ils restent justifiés au regard de l'objet du marché public. Ce cadre juridique permet de promouvoir les circuits courts pour les produits de l'agriculture, de diminuer le coût des intermédiaires

qu'il appartenait à tous les acheteurs publics de s'assurer que les procédures de passation des marchés de la restauration collective recourent aux moyens mis à disposition par le droit de la commande publique afin de favoriser l'ancrage territorial de la production,

la poursuite des tirs à balles réelles par l'armée israélienne contre les manifestants de Gaza, notamment depuis le début de la « marche du retour ». Ces tirs ont fait de nombreux morts et un très grand nombre de blessés. La diplomatie française a fait part de son inquiétude

disproportionné de la force par l'armée israélienne, les tirs mortels et mutilants par armes de guerre continuent. Des organisations non gouvernementales importantes, dont Médecins sans frontières, soupçonnent l'utilisation de munitions non conventionnelles, particulièrement mutilantes, notamment sur les membres inférieurs. Ces faits d'une extrême gravité imposent la prise de mesures d'urgence par le Gouvernement français. À ce titre, je souhaite rappeler que les territoires palestiniens, dont la bande de Gaza, sont sous occupation militaire. Israël doit dès lors, comme l'a indiqué en 2004 la Cour internationale de justice, se conformer à la quatrième convention de Genève,

si la France est prête à soutenir au plus haut niveau la constitution d'une commission internationale d'enquête, à demander la suspension de toute coopération militaire tant que la lumière n'aura pas été faite sur les tirs israéliens, à décider un embargo sur les échanges d'armes, de composants et de technologies enfin, à soutenir la procureur de la Cour pénale internationale, pour passer du stade de l'examen préliminaire à une instruction en bonne et due forme pour les crimes de guerre commis en Palestine, en particulier à Gaza. La parole

Depuis le 30 mars dernier, le bilan humain du mouvement de protestation populaire dit des « marches du retour » s'élève à près de 180 morts et 19 000 blessés, dont plus de 5 000 blessés par balles, y compris parmi la jeunesse gazaouie. Le Président de la République a exprimé, lors de ses entretiens avec Mahmoud Abbas et Benyamin Nétanyahou, sa condamnation des tirs indiscriminés des forces armées israéliennes contre les manifestants. Il a rappelé le devoir de protection des civils, en particulier des mineurs, et le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement. Il a également insisté sur la nécessité de faire en sorte que les manifestations demeurent pacifiques et a appelé tous les responsables à la retenue et à la désescalade. Il a aussi rappelé notre attachement à la sécurité d'Israël, ainsi que notre condamnation de toute forme d'incitation à la violence ou de choix politiques soutenus par certains groupes, dont le Hamas. À ce titre, la France a condamné fermement les tirs de roquettes revendiqués par le Hamas, qui ont visé Israël. S'agissant du Hamas, la position de la France est connue : ce mouvement est inscrit sur la liste des organisations reconnues comme terroristes par l'Union européenne. La position de l'Union européenne sur le Hamas ne pourra évoluer que s'il répond aux attentes bien connues de la communauté internationale. Comme vous le savez, un projet de résolution condamnant les tirs de roquettes du Hamas est en cours de discussion à New York. La France prend une part active à son élaboration, en vue de parvenir à un texte conforme à notre position. pays s'est mobilisé aux Nations unies. Il a notamment soutenu, devant l'assemblée générale, la résolution relative à la protection des civils palestiniens à Gaza, adoptée le 13 juin 2018. La France a également soutenu, lors de la session spéciale du Conseil des droits de l'homme, le 18 mai dernier, la création d'une commission d'enquête indépendante internationale chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, du droit international et du droit international humanitaire dans les territoires palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza. Un premier rapport oral a été rendu lors de la session du Conseil des droits de l'homme de septembre 2018. La commission d'enquête rendra son rapport écrit lors de la session de mars 2019. La France est par ailleurs engagée pour contribuer au règlement de la crise humanitaire que traverse la bande de Gaza. Ainsi, en 2018, nous avons financé un don de matériel à l'hôpital militaire jordanien de Gaza, ainsi que trois projets répondant à l'urgence médicale et mis en oeuvre par Médecins du monde, Humanité & Inclusion et l'UNICEF, pour un montant de plus de 650 000 euros. Au-delà, la France reste convaincue de la nécessité de parvenir à une solution politique durable à Gaza. Les conditions sont connues : la concrétisation de la réconciliation interpalestinienne et le retour complet de l'Autorité palestinienne à Gaza, d'une part, la levée du blocus israélien, d'autre part, en prenant en compte les préoccupations de sécurité d'Israël. Nous appelons donc l'ensemble des parties à prendre leurs responsabilités en ce sens. Enfin, la question de Gaza ne peut être séparée de celle du règlement du conflit israélo-palestinien dans son ensemble. À cet égard, notre pays reste pleinement engagé

Le commerce légal de l'ivoire dans l'Union européenne favorise le braconnage. C'est une évidence. En servant de couverture au commerce illicite, les exportations légales à partir de l'Union européenne contribuent à alimenter la demande dans les pays consommateurs d'Asie du Sud-Est. Notre pays a interdit le commerce d'ivoire brut et restreint le commerce d'ivoire travaillé sur son territoire par l'arrêté du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national, mais le contrôle du respect de cet arrêté est très difficile, puisqu'il établit une distinction selon que l'ivoire a été travaillé avant 1947, entre 1947 et 1990 ou plus tard. En 2017, la Commission européenne a publié un document d'orientation recommandant la suspension des réexportations d'ivoire brut. Toutefois, il apparaît que l'Union européenne devrait adopter de manière urgente une interdiction globale et juridiquement contraignante de toute importation, exportation et vente domestique d'ivoire, pour ne pas favoriser le commerce illicite, responsable de l'extinction des éléphants africains. Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir nous préciser,

vous l'avez souligné, le constat est sans appel : le braconnage continue de menacer la survie des éléphants d'Afrique. C'est choquant, intolérable, criminel ! C'est pourquoi la France est engagée, au plus haut niveau, pour la lutte contre le braconnage des éléphants et le commerce illégal de leur ivoire. Lors de la précédente conférence des parties de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction, la CITES, en septembre 2016, la France et le Luxembourg ont été les seuls pays de l'Union européenne à soutenir la demande de classement de l'éléphant d'Afrique et à interdire son commerce international, sauf dans des cas où l'importation n'est pas faite à des fins commerciales. Par ailleurs, dès janvier 2015, la France a interdit la réexportation d'ivoire brut. Un décret ministériel d'août 2016, complété par un arrêté modificatif en date du 4 mai 2017, a, de plus, interdit le commerce intérieur d'ivoire d'éléphant. Le plan d'action national pour la biodiversité, publié le 4 juillet dernier, souligne que « la France portera aux niveaux européen et international la fermeture des marchés intérieurs à l'ivoire d'éléphant ». Il s'agit de de l'action n° 63. La France considère que l'Union européenne a un rôle majeur à jouer. Le plan d'action de l'Union européenne contre le trafic d'espèces sauvages, adopté en 2016, représente un pas en avant, mais nous devons mais nous devons faire davantage, comme vous le soulignez, monsieur le sénateur. C'est pourquoi, lors du Conseil environnement du 5 mars 2018, la France et le Royaume-Uni ont appelé leurs partenaires européens à fermer leur marché d'ivoire brut. J'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises

pour l'éléphant d'Afrique, du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, géré par le secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, d'Interpol, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale des douanes.

écologique et solidaire. Madame la secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur les problèmes posés par l'application stricte de la directive-cadre sur l'eau,

2000. En application de la DCE, les décisions préfectorales conduisent trop souvent à la destruction de sites, sans étude d'impact et, le plus souvent, sans avis des conseils départementaux. Les retenues et réservoirs, les canaux et les biefs sont considérés comme zones humides selon la convention de Ramsar. Ils répondent également à la définition des zones humides dans la loi française. Pourtant, les opérations de continuité écologique se déroulent sans inventaire complet de la biodiversité de ces zones humides et, par conséquent, sans évaluation du bilan global et de l'impact sur les oiseaux, les amphibiens et les végétaux. Par ailleurs, l'énergie hydroélectrique est la plus propre et la moins coûteuse des énergies renouvelables. Considérant que 90 % des sites déjà en place ne produisent pas à l'heure actuelle, il existe donc un potentiel de croissance important. Dans une logique économique et écologique, il semble que l'équipement des sites existants serait préférable à la destruction de tous les ouvrages- moulins, forges, étangs, anciennes usines hydroélectriques ou barrages -au nom de la continuité écologique. Madame la secrétaire d'État, pensez-vous faire évoluer les pratiques pour que l'ensemble du vivant aquatique soit pris en considération dans les opérations affectant le milieu ? Comment entendez-vous simplifier la conduite des projets hydroélectriques et garantir que les nécessaires mesures de protection écologique restent proportionnées aux impacts observés

2000 établissant un cadre réglementaire pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Je tiens à vous le dire tout de suite, la conciliation des enjeux liés aux transitions écologique et énergétique est possible. C'est d'ailleurs tout l'objet des politiques publiques menées par le ministère de la transition écologique et solidaire ; c'est aussi la vision que porte la France au niveau européen. D'une part, la restauration du bon état des cours d'eau est essentielle à la reconquête de la biodiversité. D'autre part, l'hydroélectricité est une énergie renouvelable essentielle. Dans la mesure où son potentiel en France est déjà bien exploité, la priorité est donc désormais d'optimiser les installations existantes, sur le plan de la production et de la puissance de pointe. Il faut donc équiper les ouvrages de turbines aux endroits adaptés, limiter les impacts, décloisonner les rivières et restaurer des habitats naturels dans d'autres secteurs. De nombreux territoires s'y emploient avec succès, bien que la conciliation locale reste complexe à atteindre. Ainsi, le Comité national de l'eau a travaillé pendant plusieurs mois en associant toutes les parties prenantes à l'élaboration d'un plan d'action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique,

territoires. Par ailleurs, concernant la protection des zones humides, la convention de Ramsar a adopté une large définition des zones humides, comprenant notamment les marécages et les marais, les prairies humides, les tourbières, les mangroves et autres zones côtières, mais également tous les lacs

les manifestations sur la voie publique, au cours desquelles des lâchers de ballons peuvent avoir lieu, sont soumises à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. En application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, seul le préfet est compétent pour prendre un arrêté d'interdiction de lâcher de ballons, dans le cadre d'une mesure relative au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Aucun texte législatif ou réglementaire ne fonde expressément l'autorité administrative à interdire de façon générale et absolue le lâcher de ballons ni à le soumettre à un quelconque régime d'autorisation préalable. Pourtant, selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, les ballons font partie des dix déchets récréatifs le plus fréquemment retrouvés sur le littoral. Des débris de ballon sont ingérés par des dauphins, des tortues ou des oiseaux, entraînant une obstruction de leur appareil digestif, et donc leur mort inéluctable. Au mieux, ils s'accumulent sous forme de microdéchets dans les organismes de nombreuses espèces, ou polluent purement et simplement les mers. En France, les lâchers de ballons sont réglementés par certaines préfectures. Dans le département d'Ille-et-Vilaine, l'arrêté du 21 novembre 2014 les interdit dans les communes classées Natura 2000, les communes littorales et les communes particulièrement exposées aux feux de forêt, ces ballons pouvant se retrouver ensuite dans les massifs ou le milieu marin, et constituer des déchets éventuellement nocifs pour la faune et la flore. À Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Bouches-du-Rhône, les préfets ont aussi pris des mesures d'interdiction liées à des considérations environnementales. Il faut savoir que les matières plastiques représentent aujourd'hui 85 % des déchets trouvés sur les plages travers le monde. Je souhaiterais savoir si le Gouvernement entend prendre rapidement des dispositions pour préserver l'environnement, notamment dans les départements littoraux ou dans les outre-mer.

comme vous le signalez, brisant ainsi un tabou, les ballons de plastique et les fragments qui en sont issus sont une cause importante de dégradation de la biodiversité.

national et européen. La France a ainsi largement contribué à l'élaboration du projet de directive européenne sur les plastiques à usage unique, qui devrait être adopté d'ici à la fin de l'année.

Historiquement, la Lorraine doit à sa position géographique d'être, depuis l'Antiquité, un espace d'échanges et de passages entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Aujourd'hui, de nombreuses problématiques se font jour, car les réseaux de transports sont de moins en moins adaptés à l'augmentation des flux et aux mutations profondes de leur nature, conjuguée à l'impérieuse nécessité de prendre en compte la transition écologique. Si les Lorrains peuvent saluer la mise en oeuvre de la ligne à grande vitesse de Paris à Strasbourg, qui fut longtemps attendue, ils ne peuvent que s'inquiéter des récents développements intervenus dans le domaine

La suppression de la ligne ferroviaire directe entre Metz et Nice contraindra les Lorrains à passer par Paris ou Strasbourg, c'est-à-dire, souvent, à privilégier la voiture, alors que l'utilisation de ce mode de transport et son impact environnemental pouvaient

Sans résoudre pour autant ni le problème de l'encombrement de cet axe, puisque le nouveau tracé débouchera sur un entonnoir, ni la question environnementale, le Gouvernement entend le rendre payant pour tous, sans distinction entre les transporteurs poids lourds, les travailleurs transfrontaliers et les utilisateurs occasionnels. C'est une attaque supplémentaire contre le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Au total, les Lorrains ont le sentiment que le Gouvernement va à rebours de l'histoire et de la géographie de leur région, pour finalement enclaver encore un peu plus un espace territorial déjà marqué par les transformations rapides de son tissu économique. Je vous demande donc, madame la secrétaire d'État, de nous informer clairement des intentions du Gouvernement et de la SNCF quant aux suppressions de trains sur la ligne Metz-Paris, que les Lorrains ont financée, et, de manière générale, sur les mesures qu'il entend prendre afin de renforcer la position stratégique de la Lorraine au coeur de l'Europe et de permettre aux Lorrains de se déplacer librement, dans le respect de leur environnement.

fluvial « Moselle-Saône », son coût est hors de portée des financements envisageables, même avec le soutien de l'Union européenne. C'est pour cette raison que le Conseil d'orientation des infrastructures n'a pas examiné ce projet dans son rapport du 1 février 2018 et qu'il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de le relancer. Il s'agit très coûteux, à la rentabilité incertaine. Concernant ensuite la pérennité de la liaison TGV Metz-Nice, le pôle d'échanges multimodal de Lyon-Part-Dieu va connaître des travaux importants à compter de 2019, au moins jusqu'en 2023. Cette contrainte a conduit SNCF Mobilités à détourner ou à supprimer certains TGV. La liaison Metz-Nice sera ainsi interrompue en 2019. Après discussion

concernant le secteur nord du projet de l'A31 , le débat public organisé en 2015 a permis de montrer que la réalisation d'un contournement de Thionville en tracé neuf était nécessaire pour assurer la fluidité de la circulation. Cet aménagement sera réalisé de manière concomitante avec l'élargissement de l'autoroute A31. C'est afin d'exécuter ces travaux dans un délai raisonnable que le précédent gouvernement avait décidé de mettre cet axe en péage. Par ailleurs, le projet de l'A31 prend en compte les préoccupations environnementales et la nécessité de développer les solutions de transport alternatives à l'usage de la voiture individuelle. Il prévoit ainsi la mise en place d'une voie réservée aux transports en commun entre le nord de Thionville et la frontière luxembourgeoise, afin de faciliter la mise en place d'une offre de transport que l'État a récemment lancé une concertation avec le public sur le projet de l'A31 pour présenter les principales caractéristiques des aménagements envisagés et dialoguer avec l'ensemble des acteurs. Cette concertation, qui prendra fin en février 2019, est un moyen utile pour que chacun puisse faire part de son avis et de ses attentes concernant cette opération. La parole est à M.

La qualité du système électrique français a toujours été reconnue. Néanmoins, la presse spécialisée a récemment souligné, fort pertinemment, sa fragilité en période de pointe et les risques de rupture qui apparaissent actuellement. Cette situation revêt trois paradoxes. Le premier est que le risque de rupture a augmenté, malgré une baisse de la consommation essentiellement due au déclin de l'industrie. Le deuxième paradoxe est que ce risque continue d'augmenter en dépit de la mise en place de mécanismes de capacité d'effacement. Le troisième paradoxe est que les solutions les plus rapides et efficaces à mettre en oeuvre, d'un point de vue environnemental, restent marginales malgré les efforts réglementaires, d'une part, et ceux des consommateurs, notamment industriels, d'autre part. À la sortie de l'hiver 2016, lors d'un déplacement sur un site industriel en Savoie, celui de la société Ferropem, le ministre de l'industrie s'était félicité du rôle joué par l'effacement dans le système électrique. Pourtant, deux ans plus tard, les objectifs sont très loin d'être atteints.

alors même que la redevance de capacité payée par les consommateurs, dont les industriels, engendrera une ressource globale de 1,5 milliard d'euros. Pour assurer sa Pour assurer sa sécurité d'approvisionnement, la France abandonne progressivement la seule solution économique et écologique disponible dans un délai court, au profit d'outils thermiques fortement émetteurs de CO2. Leurs émissions augmentent fortement, de plus d'un million de tonnes par an. Ce choix de la France se trouve, de surcroît, à contre-courant de celui de nos voisins européens, qui mobilisent un volume d'effacement largement supérieur. C'est aussi le cas des grands États américains, dont les politiques sont plus anciennes et plus volontaristes. Lors de sa prise de fonctions, en septembre 2018, M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire a souligné à quel point, selon lui, l'écologie et l'économie pouvaient et devaient se conjuguer. Le Gouvernement est-il

La France a joué un rôle pionnier en Europe dans le développement de l'effacement de consommation. D'ailleurs, tous les marchés français de l'électricité sont aujourd'hui ouverts à la participation des effacements.

Nous disposons d'ailleurs d'un dispositif de soutien dédié à la filière, l'appel d'offres effacement, que nous avons négocié avec la Commission européenne. Cela nous a notamment permis, en 2018, de soutenir financièrement les effacements présentant les meilleurs standards environnementaux. Nous souhaitons par ailleurs améliorer encore l'attractivité de ce dispositif et le simplifier. Enfin, monsieur le sénateur, j'attire votre attention sur le dispositif d'« interruptibilité » mis en place par l'État. Il permet d'interrompre la consommation sur demande du gestionnaire de réseau de transport pour soutenir les actions des industriels concourant à la sécurité d'approvisionnement. Ainsi, monsieur le sénateur, vous pouvez constater que nous agissons sur plusieurs leviers pour permettre à la flexibilité de consommation, notamment

écologique et solidaire. Le déficit hydrique en France se chiffre en millions de mètres cubes d'eau ; il pourrait se compter en milliards, en période d'étiage, d'ici à 2050. Conséquence directe de cette carence, le rendement des vignes et des céréales chute de façon drastique. Les acteurs des filières agricoles et environnementales n'ont pas tardé à tester différentes solutions pour pallier ce manque d'eau. L'une d'elles consiste à réutiliser des eaux usées afin d'optimiser la gestion de l'eau et d'anticiper ainsi sa rareté annoncée. Si les premiers résultats semblent encourageants en termes de rendements des champs ainsi irrigués, aucun suivi des résidus médicamenteux contenus dans les rejets des stations d'épuration ayant servi à ces irrigations n'a encore été réalisé. Pourtant, un rapport émanant de l'Académie nationale de pharmacie nous alerte : « Rien dans les cahiers des charges ne spécifie aux stations d'épuration de devoir garantir l'élimination spécifique de molécules ciblées, sachant que les égouts, malheureusement encore appelés tout-à-l'égout, recueillent tout ce que les populations, les établissements de soins, les locaux industriels ou municipaux, les commerces et petites industries peuvent y déverser. » Ces eaux usées, distinctes des eaux qui sont destinées à la consommation humaine,

Dans un rapport d'étude, l'université hébraïque de Jérusalem constate qu'il y a bien migration des contaminants présents dans les eaux usées vers les plantes irriguées et que la compilation des substances chimiques en décuple les effets. Madame la secrétaire d'État, avant d'envisager de réutiliser les eaux usées provenant des stations d'épuration, sachant que celles-ci ne traitent ni les résidus médicamenteux ni bien d'autres choses encore, il est urgent d'appliquer un principe de précaution et d'interdire pour l'heure cette pratique. Ma question est la suivante quelles mesures comptez-vous prendre pour garantir l'élimination de ces substances par les usines de traitement d'eau et éviter ainsi le risque de contamination des plantes irriguées, et donc de la chaîne alimentaire ?

Les enjeux de santé et d'environnement sont au coeur de l'action du Gouvernement, qui met en oeuvre plusieurs plans et stratégies ayant vocation à réduire les pollutions par les substances chimiques. Je sais que vous les connaissez bien, madame la sénatrice : nous avons eu l'occasion d'échanger sur cette question. S'agissant des substances chimiques présentes dans les eaux usées traitées, les réglementations européennes et françaises en matière d'assainissement sont en cours de structuration. Elles prévoient que les stations de traitement des eaux usées urbaines soient conçues, dimensionnées et exploitées pour réduire la pollution organique et, le cas échéant, la pollution azotée

ainsi été demandé aux collectivités, par une note technique du 12 août 2016, de rechercher certains micropolluants dans les eaux usées traitées et dans les eaux brutes des stations de traitement, d'identifier leurs sources d'émission en amont des stations et d'engager une démarche de réduction. Lorsque les eaux usées traitées sont réutilisées pour l'irrigation des cultures ou l'arrosage des espaces verts, des exigences supplémentaires sont appliquées pour réduire la présence de micropolluants et les risques d'exposition des sols aux métaux lourds. Ces questions ont également fait l'objet de travaux spécifiques d'évaluation des risques menés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La France est l'un des cinq pays européens à réglementer la réutilisation des eaux usées traitées. Des discussions sur ce sujet sont en cours au niveau européen, sur la base d'un projet de règlement visant à homogénéiser les règles encadrant l'irrigation

Dans chaque commune, dans l'Hexagone comme dans les outre-mer, nous sommes désormais confrontés à la recrudescence d'un comportement révélateur d'un réel incivisme et particulièrement dommageable pour l'environnement. Les infractions aux règlements de collecte se multiplient.

ces comportements des problèmes en matière de sécurité, la voie publique étant encombrée, et surtout en matière de salubrité, le dépôt de déchets non réglementaires étant nocif pour l'environnement. Ainsi, à La Réunion, ces dépôts entraînent la multiplication des gîtes larvaires en période préendémique peuvent également engendrer des pollutions au plomb, et donc provoquer des cas de saturnisme. Or, pour mener la lutte contre le fléau des décharges sauvages, il apparaît que le montant des amendes forfaitaires des contraventions de la deuxième et de la troisième classe le non-respect de la réglementation en matière de gestion des déchets n'est pas suffisamment dissuasif. Il est donc urgent de se saisir du sujet en instaurant une répression plus dissuasive.

la peine d'amende maximale, soit 150 euros, au lieu de 35 euros, pour les infractions visées à l'article R. 632-1 du code pénal, et 450 euros, au lieu de 68 euros,

Ainsi, les infractions visées à l'article R. 632-1 deviendraient des contraventions de troisième classe, ce qui porterait le montant de l'amende forfaitaire à 68 euros, au lieu de 35 euros, et celles visées à l'article R.

Deuxièmement, un groupe de travail dédié a proposé des modifications législatives et réglementaires pour lutter plus efficacement contre les dépôts illégaux de déchets. Ces propositions, que nous voulons très concrètes,

nous la prenons, elle aussi, au sérieux. Troisièmement, un guide pratique visant à aider les maires à faire usage de leurs pouvoirs de police pour sanctionner l'abandon de déchets sera réalisé. Nous devons être aux côtés des collectivités territoriales et des élus locaux pour lutter contre ce fléau. Enfin, un travail spécifique est mené sur la question de la reprise à titre gratuit des déchets du bâtiment, qui constituent souvent l'une des premières sources de dépôts sauvages. Vous m'interrogez également, madame la sénatrice, sur la possibilité d'appliquer le montant maximum des amendes. C'est déjà prévu. L'agent qui constate une infraction a deux possibilités. La première est d'appliquer l'amende dite « forfaitaire » : c'est une procédure simplifiée pour les contraventions des quatre premières classes ; elle permet de sanctionner immédiatement l'infraction, en contrepartie d'un montant minoré. La seconde est d'envoyer un procès-verbal au procureur, qui le soumettra à l'appréciation du juge : dans ce cas, le contrevenant s'expose à l'amende maximale prévue.

que SNCF Réseau pourrait ne plus exploiter à l'horizon 2023 si aucune amélioration n'intervenait d'ici là. Cela serait calamiteux et insensé au vu du bassin de vie que représente Le Mans, qui alimente Alençon. Pour rappel, Pour rappel, ce n'est pas une petite ligne : elle fait partie d'un ensemble reliant quatre chefs-lieux de département et trois régions. Elle est donc essentielle au développement des territoires, mais aussi au bien-être de leurs habitants. Une demande expresse de financement d'urgence, pour un montant de 3 millions d'euros, a d'ailleurs été adressée au Gouvernement par la présidente de la région Pays de la Loire. Je vous demande donc, madame la secrétaire d'État, de garantir en toute urgence les engagements de l'État relatifs à cette ligne et, plus particulièrement, de nous indiquer expressément le calendrier de déblocage des fonds prévus en compensation de l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes. Il faut savoir que tout retard ou report de paiement, notamment au titre de 2021, comme nous avons pu l'entendre, affectera forcément de manière inquiétante le démarrage de la procédure de travaux de ce chantier. Il ne faut pas que la modernisation du réseau existant, en ce qui concerne les lignes du quotidien, et particulièrement les lignes TER, qui sont au bord de l'implosion, soit délaissée au profit de grands projets tels que le Grand Paris Express : celui-ci, on le sait, engloutira en effet, sur plusieurs dizaines d'années, bon nombre d'investissements

Les besoins de remise à niveau de ces lignes représenteront plusieurs centaines de millions d'euros d'investissements par an durant la prochaine décennie. Nous pouvons vous assurer, monsieur le sénateur, que l'État demeurera au côté des collectivités territoriales, au premier rang desquelles les régions, pour préserver ces liaisons dans le cadre des S'agissant de la ligne Caen-Alençon-Le Mans, le Gouvernement partage vos inquiétudes sur l'état des infrastructures, en particulier pour la partie de cette ligne située entre Le Mans et Alençon.

Il va de soi que l'État envisagera un effort important dans le contexte de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous nous y sommes engagés, et nous tiendrons cet engagement. Les financements correspondants, qui ne figurent pas dans le CPER actuel, seront inscrits dans le contrat d'avenir pour la région Pays de la Loire. Ce nouveau pacte en faveur des territoires ligériens entérinera les engagements de l'État à la suite du rapport de la mission sur les mobilités du Grand Ouest. Au-delà de ces travaux, il importe d'assurer la pérennité de la ligne sur le long terme. C'est dans le cadre des réflexions qui s'engagent, en partenariat avec les régions, autour de la mise en place de solutions techniques et de gouvernance novatrices et adaptées aux enjeux propres à chaque infrastructure que des réponses seront apportées pour cette ligne.

Toutefois, l'ARAFER, dans son avis 2017-049 du 14 juin 2017, a rejeté les propositions d'APRR et d'Artelia, motivant sa décision par un manque de justification des dépenses. Or, en juin dernier, l'A36 a de nouveau été lourdement inondée à hauteur de Burnhaupt-le-Bas. La préfecture du Haut-Rhin a interpellé APRR, dans un courrier en date du 17 août 2018, pour que l'entreprise lui transmette un dossier prenant en compte l'intégralité du problème lié aux inondations. La sécurité des usagers de l'autoroute est en jeu, mais également celle des habitants de Burnhaupt-le-Bas.

du fait du changement climatique. Par ailleurs, cette commune a été classée trois fois en état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. Compte tenu des déclarations de catastrophe naturelle intervenues et de la fréquence des inondations,

Pourtant, les épisodes climatiques des dernières années justifient un réaménagement profond des évacuations d'eau de l'A36 à hauteur de Burnhaupt-le-Bas. Les élus locaux font état de leur incompréhension devant un refus d'aménagement de l'autoroute A36 malgré la survenue de plusieurs inondations ces dernières années. Madame

Le 24 juillet dernier, le Conseil d'État a toutefois jugé que l'opération considérée ne pouvait pas être intégrée à ce plan d'investissement autoroutier, au motif qu'elle relevait des obligations contractuelles du concessionnaire. Cette opération a ainsi été retirée du plan, mais elle se fera dans un autre cadre juridique. Il revient en effet au concessionnaire de réaliser ces travaux d'aménagement sans compensation, conformément à ses obligations contractuelles. Je tiens à vous assurer que l'aménagement prévu sur l'autoroute A36 ne sera en rien, comme vous le craignez, un aménagement, et que la ministre sera tout particulièrement vigilante à sa bonne réalisation

avec la proposition modifiant le tracé du corridor RTE-T mer du Nord-Méditerranée, qui identifie un lien direct entre les ports irlandais, belges et néerlandais, mais en excluant les ports français. Ce texte entrer en vigueur qu'en cas de sortie « sèche » du Royaume-Uni de l'Union européenne, son examen ne débutera qu'une fois que le Parlement britannique se sera prononcé sur l'accord de retrait récemment trouvé. La France doit se préparer à la sortie du Royaume-Uni, quelles que soient ses modalités. Nous identifions et anticipons donc toutes les hypothèses. Tel est l'objet des plans de contingence que le Gouvernement a établis et du projet de loi l'habilitant à prendre par ordonnances les mesures de préparation au Brexit, notamment pour réduire les délais d'aménagement des infrastructures nécessaires dans certains ports. La préparation des ordonnances a également débuté avec l'appui du coordonnateur interministériel afin que leur contenu soit au plus près des besoins. Les services de la ministre sont en contact régulier avec les ports concernés. vous avez eu l'occasion de contribuer à ces réflexions. Concernant les financements, le Gouvernement a demandé et obtenu, lors du dernier appel à projets « transport » du mécanisme d'interconnexion en Europe, que soient bien inclus les ports.

pression pour que les ports français aient toute la place qu'ils méritent ! La ministre s'est également rendue à Dublin, le 23 novembre dernier, pour sensibiliser les autorités irlandaises aux atouts des ports français. Nous travaillons donc pour que les intérêts des ports français soient défendus dans l'immédiat et sur la période budgétaire 2021-2027, pour laquelle les négociations sont en cours. Monsieur le sénateur, merci de votre implication et de votre soutien. C'est ensemble que nous devons continuer à nous battre au niveau européen pour que les ports français aient toute la place

actuel. Plus de 2 milliards d'euros seront consacrés à la relance des petites lignes ferroviaires. C'est une excellente décision. J'insiste sur la nécessité d'améliorer la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port et, surtout, d'achever enfin la section Bedous-Canfranc

milliard d'euros sera consacré à la rénovation des routes nationales. Il est impératif que la RN 134 soit inscrite comme une priorité dans le programme de rénovation. Cet axe est aujourd'hui totalement inadapté au trafic transfrontalier et son niveau de sécurité est déplorable.

Nous parlons pourtant ici de la troisième traversée pyrénéenne ! Elle souffre de la comparaison avec la partie aragonaise et elle ne permet pas au Béarn de tisser des liens avec l'Espagne. J'ajouterai que, en termes de désengorgement de l'agglomération bordelaise, l'axe européen E7, dans sa section Pau-Langon-Limoges, constitue une alternative crédible.

Le projet de loi sur les mobilités contient de bonnes mesures, mais j'attends que vous nous rassuriez sur la réponse aux justes attentes des Basques et des Béarnais en termes d'infrastructures routières et ferroviaires et, surtout, sur le financement et le calendrier de ces investissements. La parole

En complément, 7,85 millions d'euros, dont 75 % financés par l'État, sont programmés au titre d'une enveloppe hors CPER. Entre Pau et Oloron, 11 millions d'euros vont être

en début d'année prochaine. Comme vous le savez, monsieur le sénateur, le département des Pyrénées-Atlantiques a repris à son compte un projet de voie rapide Pau-Oloron. Il est donc porté par la collectivité, qui en assume la responsabilité. S'agissant de la section comprise entre Oloron et la frontière espagnole, des travaux d'aménagement de points singuliers sont inscrits à l'actuel CPER à hauteur de 7 millions de francs, pris en charge en totalité par l'État. Les volets Les volets suivants ont été identifiés : le traitement d'aménagements physiques ponctuels, notamment les entrées nord et sud d'Asasp-Arros ; la mise en place d'équipements d'information des usagers ; la réduction de la vulnérabilité face aux aléas naturels. Les études sont en cours, pour un lancement des premiers travaux l'année prochaine. Enfin, en ce qui concerne la déviation d'Oloron-Sainte-Marie, un montant de 77 millions d'euros est inscrit à l'actuel CPER, cofinancé à parité par l'État et le département des Pyrénées-Atlantiques. La déclaration d'utilité publique de 2008 a été prorogée jusqu'en mars 2023. Les études de conception détaillée, complexes compte tenu de la nature des ouvrages à réaliser- notamment des viaducs et un tunnel -, se poursuivent, de même que les procédures préalables à l'engagement des travaux. Comme vous le signalez, monsieur le sénateur, un surcoût est en effet attendu. Il est notamment dû à des contraintes géotechniques très fortes dans le secteur. Une fois le montant de ce surcoût fiabilisé, une discussion avec les collectivités cofinanceuses sera nécessaire pour envisager les modalités de financement. En définitive, comme vous pouvez le voir, l'État est pleinement mobilisé pour aménager l'axe de la RN 134 en cohérence avec la réalité des besoins de mobilité de ce territoire que vous défendez si bien, monsieur le sénateur

avez évoquées a en effet été reportée à la fin de 2019, afin de tenir notamment compte des délais pris par les concessionnaires pour les dévoiements de réseaux. Effectués en souterrain dans un milieu urbain dense, les travaux ont nécessité de congeler les sols pour sécuriser le terrain et creuser les enceintes des stations. Si la méthode de congélation par saumure a fonctionné pour la station Aimé Césaire, elle s'est avérée insatisfaisante pour la station Mairie d'Aubervilliers, en raison de la présence d'une circulation d'eau souterraine qu'il était difficile d'identifier avant ces travaux. Les travaux de terrassement ont donc été temporairement suspendus jusqu'à ce qu'une alternative soit trouvée, la congélation utilisant de l'azote liquide. De telles difficultés techniques, inhérentes aux travaux souterrains, ont malheureusement des conséquences importantes sur les délais. La RATP a procédé, en lien avec les entreprises, à l'actualisation du calendrier : le 21 septembre dernier, elle a ainsi annoncé une mise en service en décembre 2021, soit avec près de deux ans de retard. Je sais l'impact que ces retards peuvent avoir sur le quotidien des riverains, monsieur le sénateur. Je peux vous assurer que le Gouvernement et la RATP restent particulièrement attentifs à la bonne poursuite du chantier. C'est une priorité pour le Gouvernement. Par ailleurs, la ministre des transports fait confiance à l'autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, pour étudier et mettre en oeuvre toutes les mesures destinées à pallier ce retard. Enfin, au-delà de ce projet, l'État est très attentif au développement des transports en Seine-Saint-Denis et y contribue fortement au travers du contrat de plan État-région.

Sur les 900 millions à 1 milliard d'euros de recettes attendus par le Gouvernement, la mise en oeuvre de cette disposition entraînera une hausse d'impôts de 700 millions d'euros pour la seule filière du bâtiment et des travaux publics À titre d'exemple, les 122 entreprises de travaux publics des trois départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze verront, de fait, leurs marges baisser de l'ordre de 40 % à 60 %, selon la spécificité de l'entreprise. Les conséquences seront extrêmement lourdes et nombre d'entreprises risquent de ne pas y survivre. Il est à craindre une casse sociale en termes de rémunérations des salariés, soit près de 3 000 personnes pour les trois départements que j'ai cités, voire des licenciements. Par ailleurs, l'effort de formation sera amoindri, du fait de la réduction des budgets dédiés. Une application brutale de ce changement fiscal est d'autant plus inacceptable que tous les marchés en cours de réalisation ou signés n'ont évidemment pas intégré cette nouvelle donne financière. En outre, les professionnels n'ont pas de solution alternative en termes d'engins, tous

? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice Perol-Dumont, le Gouvernement a souhaité que la fiscalité pour le gazole non routier à destination des entreprises industrielles, des travaux publics et du bâtiment soit la même que celle des particuliers C'est un effort important pour ces entreprises, nous en avons conscience, maïs nous avons relevé la taxation du gazole pour des raisons écologiques : l'objectif est de limiter sa consommation, qui conduit au réchauffement climatique et à la pollution de l'air. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de notre politique écologique, qui a plusieurs objectifs : orienter les investissements et les pratiques vers des solutions moins polluantes ; se substituer à d'autres impôts et taxes sur le travail et les entreprises, d'où la baisse des cotisations salariales et la suppression de la taxe d'habitation ; procurer les moyens de financer les investissements pour la transition écologique assurer une redistribution sociale et un accompagnement des acteurs les plus vulnérables, par exemple avec la généralisation du chèque-énergie ou la prime à la conversion des véhicules. Le Gouvernement, conscient des difficultés d'adaptation et de l'impact fort que peut avoir cette hausse de taxe pour certaines entreprises, a décidé de mettre en place un dispositif de transition. Il a ainsi proposé au Sénat d'assurer que la variation du prix puisse être répercutée dans les contrats en cours- cela répond, madame la sénatrice, à votre question précise -, de permettre la distribution et la consommation de GNR au tarif du gazole pendant les premiers mois de l'année pour fluidifier la logistique du produit, d'exonérer le secteur du transport frigorifique de la hausse de fiscalité pendant un an. Le Gouvernement étudie également la possibilité de mettre en place des dispositifs de suramortissement pour faciliter les investissements des entreprises de distribution de GNR et le renouvellement des équipements.

proposées, je crois que le Gouvernement, sur cette question comme sur beaucoup d'autres, devrait prendre la peine d'entendre, d'écouter, et revoir fondamentalement sa copie ! Je vous remercie,